Monsieur le président, La séance est reprise. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie ce jour sont consultables

Acte est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au et figurera dans l'analyse politique des scrutins. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.

des cas dans lesquels la Cour nationale du droit d'asile pourra statuer à juge unique dans un délai de cinq semaines. En effet, l'article 6 étend les audiences

les décisions prises après audience collégiale- cela devrait constituer la règle de droit commun -représentent déjà moins d'une décision sur deux.

de sanctions pénales du fait de l'entrée sans autorisation sur le territoire afin de solliciter l'asile, l'article 32 porte interdiction d'expulser un réfugié, sauf raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, et l'article 33 porte interdiction d'expulser ou de refouler un réfugié aux frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de son appartenance à un groupe social, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.

comme à la Cour nationale du droit d'asile. À nos yeux, la nécessité de recourir à la captation vidéo est la conséquence de la concentration des institutions chargées de l'instruction des demandes d'asile, à savoir l'OFPRA et la CNDA, dans la région parisienne.

Au vu de ces remarques, nous souhaitons donc que le recours à cette technique soit particulièrement encadré. Cet amendement vise également à mieux articuler le recours simultané à l'interprétariat et à la vidéo-audience, en prévoyant que l'interprète soit présent au côté du justiciable, et non auprès de la formation de jugement.

pour l'auditionner en visioconférence. Cette généralisation de la visioconférence est non seulement contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais aussi critiquée par les acteurs du contentieux, à commencer par les juges. Saisi de la question du recours à la visioconférence, le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision du 20 novembre 2003, que l'utilisation de cette méthode était conforme à la Constitution, à condition qu'elle soit subordonnée au consentement de l'étranger.

et examiner leur demande d'asile à distance, par écran interposé ... Cette disposition fait, bien entendu, l'unanimité contre elle. Ainsi, la Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Mme Adeline Hazan, estime que la généralisation du recours à la visioconférence pour les audiences sans le consentement des intéressés est inacceptable. Outre les difficultés techniques souvent constatées, la visioconférence entraîne, selon elle, une déshumanisation des débats et nuit considérablement à la qualité des échanges. Du côté des avocats, le Conseil national des barreaux estime qu'une audience se tenant par le biais de moyens de télécommunication est incompatible avec une défense de qualité, de surcroît lorsque l'oralité est déterminante pour arrêter la décision. Du côté des juges, tous ceux qui ont fait l'expérience de la visioconférence s'opposent à sa généralisation. Le syndicat de la juridiction administrative indique ainsi que ce dispositif a pour effet de mettre à distance le juge et les parties, qui ne se côtoient plus physiquement. Le principe pluriséculaire d'unité de temps et de lieu propre à tout procès se trouve dès lors mis à mal. En résumé, la dématérialisation des audiences en matière de droit d'asile nuit gravement au principe fondamental du droit à un procès équitable, et donc à notre démocratie.

d'asile. La possibilité, pour le requérant qui séjourne en France métropolitaine, de venir s'exprimer en personne devant la CNDA pour exposer ses arguments de fait et de droit est une garantie essentielle qu'il convient de conserver. La régression proposée est d'autant moins acceptable qu'elle est justifiée par des difficultés d'organisation des audiences. On ne peut accepter que des garanties procédurales soient altérées au nom de considérations pratiques. Une audience se tenant par vidéoconférence est incompatible avec une défense de qualité, de surcroît lorsque l'oralité est déterminante pour la détermination de la décision qui doit être prise. C'est pourquoi l'utilisation de la vidéoconférence doit être réservée aux seuls cas de force majeure, l'éloignement géographique rend impossible la présence physique du requérant.

ou pour le confort de certains demandeurs, cette procédure ne peut être généralisée et imposée aux principaux intéressés selon une logique purement pratique. Nombre des individus concernés ont besoin d'un contact humain pour pouvoir livrer un récit souvent douloureux

La présence de magistrats disposant d'une connaissance approfondie des procédures judiciaires françaises et étrangères constitue un apport non négligeable lors de l'examen de demandes d'asile. Il convient donc de ne pas décourager ces mobilités.

En conséquence, la mesure proposée est conforme aux prescriptions constitutionnelles et conventionnelles que la France doit observer, les garanties assurant le respect du contradictoire requises par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 2011 étant bel et bien prévues. Ces garanties sont les suivantes : une salle d'audience spécialement aménagée, ouverte au public et relevant du ministère de la justice, un déroulement de l'audience en direct et assurant la confidentialité de la transmission, le droit pour l'intéressé d'obtenir communication de l'intégralité de son dossier, la présence de l'avocat, la réalisation d'un procès-verbal ou d'un enregistrement. En outre, le bilan de la vidéo-audience mise en oeuvre par la CNDA pour les demandes d'asile outre-mer est plutôt positif. Cela nous a été confirmé lors de notre déplacement à la CNDA.

la possibilité, pour les magistrats de l'ordre judiciaire détachés à la CNDA, de présider des formations de jugement. Le projet de loi modifie l'article L. 233-5 du code de justice administrative pour aligner les modalités d'accueil des magistrats de l'ordre judiciaire au sein de la CNDA par voie du détachement sur celles qui sont applicables aux conseillers et premiers conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le même grade. Lors des auditions

d'asile, le CESEDA, pose trois conditions cumulatives : il doit s'agir d'une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. Cette troisième condition nous semble restreindre inutilement la possibilité offerte à la CNDA. Surtout, elle a pour effet de retarder le recours à ce dispositif, alors que, apporté au plus tôt, un éclairage du Conseil d'État pourrait garantir une plus grande sécurité juridique.

Le scrutin est ouvert.

deux autres sont plus problématiques : constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours -pourquoi et comment, on ne le dit pas -et rejeter les recours ne présentant aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'OFPRA- cela revient, en clair, à statuer d'ores et déjà sur l'appel.

rappelle que le président de la cour ou les présidents qu'ils désignent peuvent statuer par ordonnance motivée dans les cinq cas suivants : donner acte des désistements, rejeter un recours ne relevant pas de la compétence de la CNDA, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours, rejeter un recours entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou qui n'a pas été régularisée à l'expiration d'un délai indiqué par la CNDA -typiquement, l'introduction tardive d'un recours contentieux -, rejeter un -, rejeter un recours ne présentant aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'OFPRA. Dans ce dernier cas, l'ordonnance ne peut être prise qu'après examen de l'affaire par un rapporteur et après prise de connaissance des pièces du dossier par le requérant.

visant à prévoir que toute décision définitive de rejet d'une demande d'asile de l'OFPRA, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d'asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français.

Certains vont d'ailleurs plus loin et considèrent que tous les déboutés sont en fait des usurpateurs, n'utilisant le droit fondamental qu'est celui de demander l'asile que pour bénéficier temporairement d'un statut légal sur notre territoire, tout en sachant que, une fois déboutés, ils ne seront pas expulsés. Le syndrome du, sans doute ... J'ai eu l'occasion de le souligner lors de la discussion générale : ni l'allongement de la durée de rétention ni la délivrance

On s'offusque de la montée de l'extrême droite chez nos voisins européens, on dénonce avec emphase le refus de l'Italie d'accueillir l'dans ses ports, mais que faisons-nous ici de vraiment différent ? Nous adoptons, loi après loi, des dispositions toujours plus attentatoires aux droits fondamentaux, en faisant croire à nos concitoyens que la fermeté en la matière permettra de régler la crise migratoire. Mes chers collègues, tout

Alors que le rapporteur a rétabli à trente jours le délai de recours devant la CNDA après rejet par l'OFPRA d'une demande d'asile, il durcit drastiquement le dispositif d'OQTF. Ainsi, cet article prévoit que toute décision définitive de rejet d'une demande d'asile de l'OFPRA, le cas échéant après que la CNDA a statué, vaut obligation de quitter le territoire français, alors même que la jurisprudence de la CNDA montre qu'un certain nombre de demandeurs d'asile ont raison de persévérer dans leur démarche, car des statuts ou des protections subsidiaires sont régulièrement accordés par la CNDA dans ce cadre. les termes de l'association ELENA, « créer une catégorie d'" éloignables ", car, lorsque le demandeur d'asile persiste à vouloir faire reconnaître ses persécutions, c'est que le danger est prégnant et durable

ne seraient pas chargés exclusivement de veiller à l'application de la convention de Genève et d'évaluer les demandes d'asile, mais seraient en même temps et simultanément chargés d'apprécier la capacité de la personne à rester sur le territoire, en particulier le respect des conditions dans lesquelles elle devrait être éloignée, notamment au regard de la Convention européenne des droits de l'homme.

donc de la décision de l'OFPRA, et ce qui relève d'une problématique d'admission au séjour et d'éloignement, dont le traitement revient à l'autorité administrative, c'est-à-dire au préfet. Si l'OFPRA ou la CNDA devaient se prononcer sur le droit au séjour, cela les amènerait à traiter d'une multitude de questions nouvelles, liées par exemple à l'existence d'une menace pour l'ordre public ou au droit de l'étranger à mener une vie familiale normale, distinctes de leur office actuel. La modification introduite par le Sénat n'aurait donc de sens qu'avec une réforme profonde des structures chargées de l'asile et de l'immigration, qui n'est pas dans les objectifs du Gouvernement. Se poserait en outre la question du régime contentieux des OQTF, qui doivent pouvoir faire l'objet d'un recours suspensif. Or il n'est ni souhaitable ni opportun

de manière exclusive à l'OFPRA et, le cas échéant, à la CNDA -et l'appréciation du droit au séjour, qui relève d'abord de l'autorité préfectorale. Il y a ici deux régimes juridiques distincts, l'asile et le séjour : ce n'est pas parce qu'une personne ne relève pas du premier qu'elle ne peut faire une demande au titre du second. Or le dispositif introduit par la commission l'interdit. La préfecture reçoit les demandes et délivre des autorisations provisoires de séjour. Donner à l'OFPRA ou à la CNDA la capacité de délivrer une OQTF risquerait d'entraîner un imbroglio juridique. À partir du moment où un demandeur d'asile est débouté, il est évident qu'il ne doit pas se maintenir sur le territoire, mais cet article mélange les rôles des institutions qui participent à la procédure. Enfin, s'il n'y a aucune objection de principe à ce que le législateur intervienne pour modifier le partage des compétences entre les préfets et l'OFPRA,

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

l'échec des procédures de relocalisation et de réinstallation, doit-on continuer de laisser les « dublinés » errer de pays en pays ?

que l'Italie leur accordera la protection qu'ils réclament et à laquelle ils ont droit ? Non ! La France, fidèle à sa tradition humaniste, doit montrer l'exemple. Adopter notre proposition permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes, sans pour autant créer un appel d'air, pour la bonne et simple raison

Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. » Monsieur le ministre d'État, vous ne

et non par des mesures unilatérales, qui ne manqueraient pas d'avoir de très nombreux effets pervers sur le volume de la demande d'asile en France. Les clandestins sont nombreux dans notre pays à ne pas avoir fait de demande d'asile. Décider, pour le seul territoire français,

socialiste, que la France a accepté, voilà quelques années, un objectif en matière de relocalisation des demandeurs d'asile, pour soulager les pays sur les territoires desquels ils arrivaient par centaines de milliers. L'objectif était d'ailleurs bien modeste, puisque, sur les 160 000 relocalisations acceptées au niveau de l'Union européenne, la France, généreusement, a proposé la relocalisation de 6 000 demandeurs d'asile. Et encore cet objectif a-t-il rapidement paru nettement excessif

qui présiderait à certaines réponses. Je voudrais lui dire et vous dire, à vous mes chers collègues qui vous êtes exprimés

La générosité semble vous revenir maintenant que vous n'avez plus à en assumer les conséquences. Eh bien, moi, je vous le dis : responsable un jour, responsable toujours ! Oh ! Revenez sur les chemins de la responsabilité. C'est ainsi, sans doute, que vous pourrez reconquérir une certaine crédibilité.

même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des articles fixés dans le présent règlement. » Et l'article L. 742-1 du CESEDA, relatif à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile, précise : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne

les termes de l'article 17, qui vise la possibilité, pour un État, d'examiner une demande individuelle d'asile.

Il s'agit de permettre à ceux qui ne sont pas demandeurs d'asile dans un autre pays de l'Union et qui sont entrés ailleurs qu'en France de déposer leur demande en France. Ce n'est en aucune façon une régularisation générale. C'est une opportunité donnée individuellement à chaque personne entrée en Europe, ailleurs qu'en France, de demander sa régularisation dans notre pays. Ce n'est en rien une procédure qui nie l'individualisation de la demande d'asile. Je le répète, c'est une opportunité qui est donnée

des réfugiés et des demandeurs d'asile que celle que, parfois, notre jeunesse observe sur le terrain, sans comprendre où est l'idéal de notre République. Il nous a été opposé

J'essaye d'expliquer, avec mesure, que cette formulation entraîne, pour les autorités françaises, l'obligation de soumettre à l'OFPRA toute demande d'asile d'une personne présente sur le territoire qui leur sera présentée.

Le scrutin est ouvert.

des conditions dans lesquelles nous sommes contraints, en Guyane, d'accueillir ces personnes, et ce depuis de très nombreuses années. L'augmentation rapide des demandes depuis 2015 a d'ailleurs saturé le dispositif d'accueil en place. d'abord, les demandeurs d'asile se retrouvent confrontés au manque de capacités d'hébergement : aucun centre d'accueil de demandeurs d'asile de type CADA n'existe à Cayenne,

Certains demandeurs deviennent alors des squatteurs, lorsque les autres errent dans la rue au gré des opportunités. Et les squats, on les retrouve dans les anciens immeubles désaffectés de l'État, des collectivités et, même, dans le domaine privé. Autre problème,

sur des moyens en interprétariat déjà réduits. Les interprètes attendent ainsi souvent deux, voire trois ans, avant d'être payés. Je reste donc soucieux des conditions d'accueil des demandeurs d'asile, alors même que les délais d'instruction se voient accélérés. D'une part, le schéma territorial d'hébergement sera, selon toute vraisemblance, inopérant pour la Guyane. D'autre part, le manque d'hébergement reste patent et n'est pas sans incidence sur la prolifération de l'habitat informel. Je proposerai donc qu'une représentation des territoires ultramarins soit assurée au sein du conseil d'administration de l'OFII, de manière à avoir un regard avisé sur tous ces aspects.

Si bien que, dans les territoires particulièrement exposés à une pression migratoire spécifique liée à leur situation géopolitique, les structures concernées fonctionnent presque comme des centres de rétention à ciel ouvert, parce qu'il n'y a pas de solidarité entre l'outre-mer et l'Hexagone.

Houllegatte. Cet amendement a pour objet de faciliter le travail de l'interprète. En effet l'article L. 733-1-1 du CESEDA précise que les débats devant la Cour nationale du droit d'asile ont lieu en audience publique, après lecture du rapport par le rapporteur. Il est tout simplement proposé de prévoir la transmission préalable dudit rapport à l'interprète, selon des modalités qui seront fixées par décret.

Cet amendement vise à supprimer la condition selon laquelle un défaut d'interprétariat devra être imputable à l'OFPRA pour justifier du renvoi d'un examen d'une demande d'asile de la CNDA à l'OFPRA. Cette condition est un élément supplémentaire qui fige le choix de la langue. Tout le monde le sait, l'interprétariat est la seule clé pour que le demandeur d'asile ait une chance de faire entendre son récit et son parcours,

supprimer la possibilité d'entendre le demandeur dans une langue dont, je cite, « il est raisonnable de penser qu'il la comprend », dans le cas où la CNDA « ne peut désigner un interprète dans la langue demandée ». Voilà une disposition qui n'est pas acceptable au vu des enjeux.

Il est ainsi prévu de contraindre les familles à déposer une demande d'asile pour l'ensemble de ses membres. Actuellement, cet article dispose seulement que « tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'État responsable ». S'agissant des mineurs accompagnés de leurs parents, on distingue aujourd'hui deux cas de figure soit le motif de la demande d'asile repose sur les parents, et, dans ce cas, il n'y a pas de demande individuelle déposée au nom de l'enfant, mais celui-ci bénéficie, sous certaines conditions, d'un droit de séjour équivalent à celui du parent protégé parent protégé ; soit le motif de la demande repose sur l'enfant, essentiellement pour un risque de mariage forcé ou de mutilation génitale, ce qui donne lieu à une demande propre. Manifestement, ce nouvel alinéa tend à réduire le nombre de demandes d'asile en évitant la multiplication des demandes au sein de chaque famille. Or le droit d'asile est un droit individuel et non familial, sans que cela fasse ensuite obstacle à l'exercice du droit de mener une vie familiale normale de l'étranger protégé, grâce au mécanisme de réunification familiale. Ce rapprochement instille une confusion de nature à en entretenir une autre, celle qui existe actuellement entre les demandeurs d'asile et les migrants économiques. En outre, la rédaction actuelle est ambiguë et pourrait être interprétée comme occultant les cas de figure où le motif légitime de la demande repose sur l'enfant. Un examen unique de la demande d'asile d'une famille pourrait ainsi paradoxalement aboutir à une moindre protection des enfants, donc de l'ensemble de leur famille. D'autres pays, comme la Suède, prévoient justement explicitement un droit des enfants à solliciter personnellement l'asile. C'est pourquoi nous proposons de nous en tenir au droit en vigueur, faute d'une meilleure rédaction. Très bien ! Ce point précis souligne la tension qui peut exister entre le droit de mener une vie familiale normale et l'intérêt supérieur de l'enfant.

prévoyant qu'une décision de l'OFPRA n'est pas opposable au mineur lorsque la personne qui a formulé la demande n'était pas en droit de le faire. Le dispositif prévu par l'alinéa 5 de cet article est intéressant. D'une part, il offre la protection la plus étendue aux enfants mineurs. D'autre part, il établit un mécanisme protecteur lorsque la personne présentant une demande d'asile au nom de l'enfant mineur n'était, en réalité, pas en droit de le faire. Néanmoins, en l'état, la dernière phrase de cet alinéa soulève un vrai problème. En effet, la charge de la preuve repose sur l'enfant mineur qui devrait prouver que la personne présentant la demande d'asile en son nom n'est pas en droit de le faire.

de protection au titre du statut de réfugié, leurs enfants mineurs bénéficient d'une protection de même niveau.

Il n'est aujourd'hui pas tolérable que des réfugiés auxquels le droit d'asile a été reconnu dorment à la rue. Les dispositions de cet amendement ne suffiront peut-être pas à éviter les situations de rue, mais elles sont une première étape et elles s'inscrivent dans la logique de la circulaire du 4 décembre 2017.

Le projet de loi prévoit que le demandeur d'asile devra désormais indiquer dès l'enregistrement de sa demande d'asile la langue dans laquelle il préfère être entendu. Ce choix lui sera opposable pendant toute la durée de l'examen de sa demande. Cependant l'article 7 est imprécis et n'indique pas à partir de quelle étape de la procédure s'applique la règle selon laquelle le demandeur est entendu dans la langue qu'il a indiquée lors de l'enregistrement. Cet amendement vise à prévoir explicitement que le demandeur pourra introduire sa demande devant l'office soit en français, soit dans la langue qu'il aura indiquée lors de l'enregistrement de sa demande. Actuellement, l'article R. 723-1 oblige le demandeur à déposer sa demande d'asile « en français sur un imprimé établi par l'office ». Or obliger des demandeurs d'asile qui, dans la très grande majorité des cas, ne maîtrisent pas notre langue à rédiger en français les motivations de leur demande est une absurdité. Face à cette obligation, les demandeurs d'asile se trouvent souvent démunis, ce qui fait notamment le jeu des trafics de traduction. De prétendus traducteurs, contre rémunération, fournissent aux demandeurs des récits « clés en main » en français.

Alors même qu'ils justifieraient d'un dossier solide leur permettant de bénéficier d'une protection, ils se trouvent prisonniers d'un récit fabriqué de toutes pièces qui va d'emblée les décrédibiliser.

L'article 7 du projet de loi dispose que le choix de la langue de la procédure est prévu dès l'enregistrement de la demande d'asile à la préfecture. Il est ensuite opposable pour l'entretien personnel à l'OFPRA et lors du recours devant la Cour le dépôt de la demande d'asile à l'OFPRA doit toujours se faire en français. Cela peut interroger, dans le contexte du droit d'asile où les personnes sont en grande majorité non francophones. Toutefois, conformément à l'article 2 de la Constitution selon lequel « la langue de la République est le français », l'usage du français est imposé aux usagers, que sont les demandeurs d'asile, dans leurs relations avec les administrations. Des dispositions qui reconnaîtraient un droit à pratiquer une autre langue que le français dans la vie publique seraient contraires à la Constitution. En conséquence, les problématiques que vous soulevez, qui sont bien réelles, ne peuvent trouver de réponse que dans l'assistance des demandeurs d'asile

c'est bien le demandeur d'asile qui se trouve pénalisé et qui n'est pas en situation de défendre sa demande.

Or la nouvelle formulation retenue par le projet de loi, à savoir « dans une langue dont il a une connaissance suffisante », laisse supposer que l'on pourrait se contenter d'une simple connaissance d'une langue, sans s'assurer que le demandeur d'asile la comprend réellement. En En outre, le demandeur doit opérer un premier choix linguistique lors de l'enregistrement de sa demande, qui lui sera opposable durant toute la durée d'examen de la procédure, y compris en cas de recours devant la CNDA. Nous estimons, comme l'a également souligné la Commission nationale consultative des droits de l'homme, que la rigidité de ce dispositif est un frein à l'équité de l'ensemble de la procédure d'asile.

Or tout justiciable a le droit d'être entendu dans une langue qu'il maîtrise ou dont il aurait une connaissance suffisante pour comprendre et être entendu. Le sens de notre amendement est de rétablir ce droit, qui devrait être sacralisé. N'oublions pas la situation de ces exilés, qui jouent bien souvent leur vie lorsqu'ils motivent leur demande d'asile.

Le projet de loi prévoit la détermination du choix de la langue au stade de l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cadre de l'instruction de la demande d'asile devant l'OFPRA et la CNDA, le demandeur d'asile n'est pas seulement informé de ses droits : il a vocation à faire valoir les arguments au soutien de sa demande par l'exposé des persécutions subies, de son histoire et de son parcours migratoire. Il importe donc qu'il comprenne les informations qui lui sont communiquées, mais aussi qu'il puisse se faire comprendre. L'amendement

Eu égard à l'importance que revêt l'entretien devant l'Office, il n'y a pas lieu d'empêcher un demandeur d'asile de bonne foi de solliciter que la procédure s'opère dans la langue de son choix. Le texte prévoit que le changement de langue est possible à tout instant s'il s'agit de procéder à l'entretien en français. Rien ne justifie, hormis des questions d'organisation interne à l'Office, que ce principe ne s'applique pas à tout changement de langue, de telle sorte que l'intéressé puisse s'exprimer au mieux et défendre son dossier.

nous avons pris conscience de l'importance du rôle des interprètes auprès de l'OFPRA et de la CNDA. De leur capacité à restituer le plus fidèlement possible le récit du demandeur d'asile dépend en grande partie la décision rendue. Nous avons été ainsi frappés de constater que, actuellement, le niveau de qualification attendu pour exercer en tant qu'interprète auprès de ces instances est fixé par l'OFPRA et la CNDA eux-mêmes.

observables, il serait pertinent de réfléchir à la création d'un corps d'interprètes spécialisés, qui disposerait également d'une formation géopolitique et juridique adaptée à cette mission bien particulière. Dans l'attente d'une telle évolution, il est proposé que le

pour réaliser les traductions nécessaires lors des entretiens. Dans le cadre de ces marchés, les interprètes doivent satisfaire aux conditions suivantes : premièrement, posséder les diplômes universitaires requis ; deuxièmement, avoir une expérience préalable en traduction ou en interprétariat maîtriser le français et une ou plusieurs langues parlées dans les pays d'origine des demandeurs d'asile ; quatrièmement, acquérir des connaissances géopolitiques, administratives et juridiques sur les pays d'origine concernés.

En l'état actuel des textes, tant les forces de sécurité que les officiers de police judiciaire se heurtent à une carence importante en interprètes agréés. Cette déficience, voire cette absence totale d'interprètes, se rencontre notamment pour le kunama, dialecte revendiqué par des migrants de la Corne de l'Afrique- Érythréens ou Éthiopiens -, l'oromo, le woilotte, le tigrinya, l'amharique ou encore le konso.

Les procédures de notification des droits dans le cadre d'une garde à vue, d'audiences ou d'auditions sont rendues difficiles, voire impossibles ; de fait, elles sont Les procédures s'interrompent. Ce sont des personnes que l'on remet à la rue, sans autre forme de procès et sans suivi. Dans un souci d'amélioration substantielle et d'efficacité des agents de l'État chargés du traitement des dossiers,

Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à assurer au demandeur faisant l'objet d'une procédure « Dublin » qu'il sera informé de ses droits et obligations dans une langue qu'il comprend.

ainsi rédigé : « Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours, ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

l'amendement n° 400 est-il maintenu ? Avant de prendre ma décision, je voudrais vous apporter un nouveau témoignage : le 26 mai dernier, sur le parking d'un supermarché calaisien, trois policiers en patrouille ont été agressés par une quinzaine de migrants.

était suspecté d'avoir porté les coups contre la jeune femme a gardé le silence lors de son audition. Les fonctionnaires de police parviendront tout de même à connaître sa langue : il s'agit du konso, un dialecte parlé par 300 personnes en Érythrée. En dépit d'une vidéo de l'agression transmise au tribunal, les policiers ont dû relâcher le migrant, en raison de l'absence d'interprète agréé au tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.

Mes chers collègues, vous ne pouvez que le constater, ce projet de loi est totalement déséquilibré. Les bonnes nouvelles étaient si rares dans le texte transmis au Sénat

C'était le cas notamment de l'article 7 , qui proposait la suppression d'une disposition de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 dite « Warsmann », à laquelle notre groupe s'est opposé il y a quelques mois, fixait à sept jours le délai de contestation devant le juge administratif d'une décision de transfert vers un autre État membre de l'Union européenne d'un étranger faisant l'objet d'une procédure Dublin. Le présent amendement tend à augmenter ledit délai pour formuler la contestation et à le rétablir à quinze jours, soit le délai qui était appliqué antérieurement à la loi du 20 mars 2018. Sans être révolutionnaire, cet article allait dans le bon sens. Nous demandons donc qu'il soit réintroduit dans le projet de loi sous sa forme initiale. La n° 228 rectifié . Cet amendement vise à rétablir à quinze jours le délai de contestation devant le juge administratif d'une décision de transfert vers un autre État membre de l'Union européenne d'un étranger faisant l'objet d'une procédure Dublin. La réduction de ce délai à sept jours, opérée par le Sénat en première lecture de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d'asile européen, est sans fondement. La parole est

Cet amendement vise à allonger les délais de recours pour les demandeurs d'asile concernés par une procédure dite « Dublin ». L'objectif qui le sous-tend est de souligner le caractère très dérogatoire des dispositions applicables aux étrangers en France, en particulier s'agissant des délais de recours. Il convient notamment de rappeler que, en droit administratif, le délai de recours de droit commun est de deux mois. Pour remettre les choses en perspective, je voudrais rappeler automobiliste, même de mauvaise foi, dispose de deux mois pour contester un retrait de points de permis de conduire. De la même manière, un voisin, même mal intentionné, dispose d'un délai de deux mois pour contester un permis de construire. Dans le droit parallèle des étrangers en France, les demandeurs d'asile visés par une procédure Dublin, même s'ils sont de bonne foi, disposent seulement de sept jours pour contester devant le juge administratif une décision de transfert vers un autre État membre de l'Union européenne, alors même que les fondements du règlement de Dublin sont aujourd'hui largement contestés. Le présent amendement vise simplement le doublement de ce délai à quinze jours, ce qui reste une durée particulièrement dérogatoire, conformément à l'engagement pris par les députés de La République En Marche lors de l'adoption conforme de la loi Warsmann.

l'Assemblée nationale a votées voilà deux mois. Elles sont entrées en vigueur. Le Conseil constitutionnel a rendu une décision : ces dispositions sont conformes à la Constitution.

Il dispose, par ailleurs, d'un délai de sept jours pour faire un recours. Tout cela a été accepté unanimement par chacune des deux assemblées.

à ne pas avoir maintenu la position qu'il défendait voilà quelques semaines. On peut s'interroger sur la continuité de la politique migratoire quand elle oscille à ce point dans un délai aussi court

Assassi, sur l'article. L'article 8 prévoit que le droit au maintien sur le territoire cesse dès la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, et non plus à partir de la notification de la décision. Cette disposition va à l'encontre de la notion de « notification », qui impose un envoi, mais aussi une réception dont il faut attester. Rappelons que, actuellement, la décision de la CNDA prend effet après sa notification au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. La mesure l'article 8 contrevient au droit à un recours effectif. Elle permettrait l'expulsion d'un demandeur alors même qu'il n'aurait eu connaissance ni du sens de la décision ni du contenu de sa motivation, et qu'il serait dès lors dans l'impossibilité de former un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois qui lui est imparti. En outre, l'article 8 prévoit d'élargir les cas où le recours devant la CNDA ne présentera plus de caractère automatiquement suspensif de l'éloignement. Seront ainsi concernés les demandeurs d'asile provenant d'un pays sûr, les demandeurs d'asile en procédure de réexamen et les demandeurs d'asile présentant une menace grave pour l'ordre public. Dans ces hypothèses, le droit au maintien sur le territoire jusqu'à la décision de la CNDA sera supprimé. Le demandeur devra saisir le tribunal administratif pour solliciter la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre jusqu'à la décision de la CNDA. Cela obligera les juges administratifs à statuer sur le fond des demandes d'asile, une compétence jusqu'à présent réservée à la CNDA. Le juge administratif devrait alors examiner les éléments sérieux de la demande d'asile de nature à justifier le maintien ou non du demandeur sur le territoire français durant l'examen de celle-ci.

et présente le risque que les deux procédures débouchent sur des décisions contradictoires. Enfin, dans une lettre adressée aux députés français et publiée le 12 mars 2018, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe s'est lui-même dit inquiet de la suppression du caractère automatiquement suspensif des recours déposés devant la CNDA par certaines catégories de demandeurs d'asile. La parole est L'objectif de toute procédure d'asile consiste à protéger une personne contre tout renvoi dans son pays, dès lors qu'il existe un risque raisonnable qu'elle soit exposée à des persécutions. La procédure d'asile constitue donc le moyen principal pour s'assurer du respect du principe de non-refoulement, ce qui interdit de renvoyer une personne sur le territoire où sa vie, sa sécurité ou sa liberté seraient menacées. Pour ne pas être théorique et inefficace, une procédure d'asile doit donc garantir que les demandeurs d'asile ne soient pas renvoyés dans leur pays, tant qu'une décision définitive n'est pas prise sur leur demande de protection. Les États peuvent établir des procédures accélérées d'examen des demandes d'asile, en veillant toutefois à ce que tous les demandeurs bénéficient des mêmes garanties procédurales, ce qui implique la possibilité de saisir une juridiction contre la décision de refus d'octroi d'une protection internationale

la CNDA, juridiction administrative spécialisée dont la mission consiste, entre autres, à reconnaître la qualité de réfugié ou à attribuer le bénéfice de la protection subsidiaire, est compétente pour examiner les demandes de protection au titre de l'asile, puisqu'elle dispose d'une compétence de plein contentieux. Le juge administratif, quant à lui, n'est le juge ni de la qualité de réfugié, définie par la Convention de 1951, ni de la protection subsidiaire, définie par la loi française. Par ailleurs, comme l'a indiqué le Conseil d'État dans son avis, le dispositif envisagé par le Gouvernement présente le grave inconvénient de multiplier les risques de discordance entre deux juridictions administratives, obligeant le tribunal administratif à porter une appréciation à laquelle il est mal préparé, et qui relève en réalité de l'offre du juge de l'asile, et ce, avant même que la CNDA ne statue. Dès lors, il est nécessaire de renoncer à cette disposition, qui est contraire aux exigences d'une bonne administration de la justice.

du droit d'asile, principe à valeur constitutionnelle, implique, d'une manière générale, que l'étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Il va sans dire que le présent article 8, qui supprime le caractère suspensif du recours devant la CNDA des décisions prises par l'OFPRA en procédure accélérée pour les demandes de ressortissants de pays d'origine sûrs et de ceux présentant une menace grave pour l'ordre public, est une atteinte sérieuse tant à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qu'à l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit effectif au recours. L'objet unique du présent article est de rendre plus facile, et surtout plus rapide, l'expulsion des demandeurs d'asile concernés. Cette disposition portera ainsi atteinte au principe d'égalité de traitement des recours et au droit à un un recours effectif des demandeurs d'asile, dans la mesure où elle permettrait leur expulsion, alors même que le recours serait toujours pendant devant la CNDA. Cet article est inconstitutionnel, parce qu'il ne respecte pas nos engagements internationaux et parce qu'il est injuste pour les demandeurs d'asile. Les auteurs du présent amendement en demandent donc la suppression.

qui a reçu une réponse négative de l'OFPRA et qui dépose un recours auprès de la CNDA n'aurait plus la possibilité, si nous adoptons cet article, de se maintenir sur le territoire. Cette disposition, qui existait avant 2015, avait déjà été censurée par la Cour européenne des droits de l'homme le 2 février 2012, dans un arrêt bien connu, contre la France.

Aussi, il a construit une usine à gaz : on demande aux tribunaux administratifs de se prononcer sur la possibilité du demandeur de rester sur le territoire, alors même que la procédure de demande d'asile n'est pas terminée.

une nouvelle dérogation au droit commun introduite dans le droit des étrangers. Il importe de rappeler que l'effet suspensif est une protection pour la personne dont la demande a été rejetée par l'OFPRA, mais également pour l'autorité susceptible de mettre en cause le droit au maintien sur le sol français : l'effet suspensif la prémunit prémunit contre le risque de mettre en oeuvre un éloignement qui serait ensuite contredit par une décision favorable de la CNDA, et garantit donc la sécurité juridique de ses actes. C'est pourquoi nous proposons de maintenir le droit en vigueur.